de demeurer, en application de la loi, maire de cette ville qui vous est tout, qui vous est chère, Marseille. Celui qui n'a pas traversé Marseille dans la voiture de Jean-Claude Gaudin, fenêtres baissées,

préside aujourd'hui la séance pour la dernière fois. Je ne m'attendais pas, monsieur le président, à votre rappel au règlement. Aussi, je ne peux m'empêcher de vous dire toute la joie, le bonheur, l'honneur que j'ai eus d'être parmi vous. Au moment où les hommes et les femmes engagés dans la vie publique sont si injustement critiqués, je suis fier d'avoir été parmi vous. Beaucoup, auprès des ministres, ou les ministres eux-mêmes, ont eu la chance de faire de grandes écoles et d'obtenir de nombreux titres universitaires. Ici, nous sommes nombreux à avoir suivi un autre parcours, avoir gravi un à un les échelons de notre vie démocratique. C'est vrai ! Ici, nous avons reçu souvent, les uns et les autres, le sacrement du suffrage universel. Ici, et c'est mon cas, nous avons appris le droit constitutionnel et, plus encore, le respect, la considération du parcours politique de chacun.

j'ai pour vous tous un immense respect, et beaucoup d'amitié. Je ne résiste pas, en cette occasion, à la tentation de vous le dire : vous êtes des élus exemplaires de la République.

Cette mesure fait l'unanimité contre elle : les bailleurs considèrent qu'il s'agit d'un emplâtre sur une jambe de bois et toutes les associations étudiantes, y compris l'UNI, la dénoncent, ainsi que les associations pour le droit au logement et les syndicats. Non, cinq euros, ce n'est pas de l'argent de poche, contrairement à ce qu'affirment certains députés du groupe La République en Marche. C'est malheureusement le reste à vivre pour trop de familles. C'est l'argent nécessaire pour acheter le pain et les aliments de base. Sur l'année, cela représente soixante euros, soit l'équivalent d'un caddie de courses hebdomadaires. Cinq euros, c'est aussi deux jours de cantine pour un enfant.

Le Gouvernement fait les poches aux pauvres, alors qu'il s'apprête, en supprimant la part immobilière de l'impôt sur la fortune, à faire un nouveau cadeau de 3 milliards d'euros aux Français les plus riches. Cherchez l'erreur ! Ne nous parlez pas d'économies : 400 millions d'euros par an, ce sont des économies de bouts de chandelle Nous avons des propositions autrement plus justes et plus efficaces : attaquez-vous, par exemple, à l'évasion fiscale qui coûte chaque année 80 milliards d'euros à l'État ; instituez une véritable taxe sur les transactions financières qui rapporterait 36 milliards d'euros par an attaquez-vous au logement cher et aux salaires trop bas. Nous savons tous que ce n'est pas en baissant les APL que nous ferons baisser les loyers. Au contraire, c'est en construisant plus de logements, par le biais d'aides à la pierre à la hauteur et en régulant les prix du logement, que nous y parviendrons. L'État doit protéger les plus faibles, les plus fragiles, et garantir à tous l'accès aux droits essentiels. Vos décisions sont une véritable marche arrière. Nous vous demandons donc de renoncer à cette mesure anti-pauvres et anti-jeunes, indigne de notre République, qui ne devrait oublier personne. Mon cher je vous donne acte de votre déclaration. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Le décret-loi de novembre 1939, destiné à permettre la perception de cette « contribution », était clairement justifié par les circonstances de guerre. L'impôt fut d'ailleurs assorti d'une contribution exceptionnelle- sans doute pour tenir compte des circonstances -que le gouvernement de l'État français s'empressera de supprimer à l'été 1940, une fois consommées la défaite et la honte d'un armistice réduisant les effectifs de l'armée française Les esprits chagrins auront d'ailleurs remarqué que le « stoppage » ne concernait que les revenus aisément repérables et contrôlables et nullement ceux du capital ou du patrimoine. Le dispositif disparut en 1948 pour faire place au célèbre « impôt sur le revenu des personnes physiques » unifiant impôt cédulaire d'antan et progressivité pour les revenus plus importants. Chacun sait toutefois que les trente dernières années de notre histoire fiscale ont été marquées par des coups de rabot successifs sur la progressivité de l'impôt, avec notamment la suppression de l'abattement de 20 % sur les traitements et salaires, et par la montée en puissance d'un autre impôt sur le revenu, à caractère proportionnel, à savoir la contribution sociale généralisée. La CSG, aujourd'hui, rapporte davantage que l'impôt progressif, et rapportera plus encore avec la ponction supplémentaire liée au basculement des cotisations chômage et de la cotisation maladie résiduelle. La retenue à la source de l'impôt sur le revenu doit donc clairement être regardée comme la première étape vers la fusion-confusion entre impôt sur le revenu et contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, vers l'étatisation renforcée de la sécurité sociale. C'est précisément ce dont nous ne voulons à aucun prix. Rappelons enfin que la retenue à la source n'est pas la panacée contre la fraude fiscale : des pays comme l'Italie ou la Grèce la pratiquent de longue date.

Alors que les entreprises croulent déjà sous les obligations administratives, on envisage de les charger d'une nouvelle tâche, celle de prélever l'impôt sur les salaires.

C'est pourquoi nous avons confié une étude à un cabinet indépendant afin d'évaluer l'impact, pour les entreprises, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Les résultats de cette étude accessible en ligne sont frappants ; ils ont été rappelés, d'ailleurs, par le rapporteur général de notre La mesure aurait un coût initial d'environ 1,2 milliard d'euros la première année, et un coût récurrent de l'ordre de 100 millions d'euros. Plus grave encore, 75 % du coût total de la mesure serait assumé par les TPE de moins de 10 employés. Au-delà de la question du coût, l'étude montre que les chefs d'entreprise craignent une dégradation des relations sociales, en raison de l'immixtion des entreprises dans la vie privée des salariés. Ils redoutent également l'apparition de revendications salariales liées à la diminution de la rémunération nette figurant sur le bulletin de paie. Ces éléments sont à prendre en compte au moment où l'on souhaite favoriser le dialogue social au sein des entreprises ! C'est le rôle de la délégation aux entreprises de vous alerter sur ces risques, monsieur le ministre, et nous nous réjouissons de l'évolution du texte résultant des travaux de nos collègues de la commission des finances et de la commission des affaires sociales. de son amendement n° 152, le Gouvernement explique qu'il n'aura pas le temps de tester le prélèvement mensualisé et contemporain ; un tel dispositif permettrait pourtant de corréler instantanément revenu et impôt sans que les entreprises portent le poids du dispositif. La France souffre de trop nombreuses réformes menées sans étude d'impact préalable sérieuse ; nous ne cessons, après coup, de légiférer pour réparer des erreurs qu'une évaluation aurait permis d'éviter. Ne commettons pas, une nouvelle fois, une telle erreur collective

Je rappellerai simplement que ce prélèvement est une mesure de justice pour les contribuables qui voient leur situation fiscale évoluer d'une année sur l'autre. Ce n'est pas marginal : 30 % des contribuables français sont concernés chaque année. En rendant le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus et en évitant le décalage d'un an, cette mesure protège ceux qui subissent une perte de revenus de manière parfois choisie, mais parfois subie. Le paiement est également mieux réparti, puisque l'impôt sera prélevé sur douze mois au lieu de dix.

Par ailleurs, la commission des finances, sur l'initiative de son rapporteur général, dont la démarche est logique, a complété l'article 9 par certaines dispositions auxquelles nous ne sommes pas favorables, s'agissant notamment de la réduction de la charge induite pour le tiers collecteur. tiers collecteurs, il y en a déjà pour la TVA ! Je rappelle que le prélèvement à la source représente une ligne de plus à remplir sur la déclaration sociale nominative, la DSN, vaste chantier

Bien sûr, dans la ville que vous aimez et défendez avec talent, nous eûmes des orages ! On ne traverse pas quarante ans de combats et de batailles politiques sans nuages ni tensions. Mais ces affrontements étaient destinés à faire plus et mieux pour Marseille, ce qui nous a permis, monsieur le président, de surmonter toutes les tempêtes, même les plus terribles Vous manquerez à la Haute Assemblée, mais, pour ma part, j'ai l'assurance-et j'aurai la chance -de vous retrouver dans quelques jours, ou quelques heures, sous la protection de la Vierge de la Garde, ... Priez pour nous ! ... qui vous accompagnera encore longtemps. D'autres piaffent pour vous succéder ; je sais qu'avec votre intelligence et votre sens des responsabilités, vous saurez vous garder de vos amis comme de vos ennemis. Merci pour tout, cher Jean-Claude Gaudin

de préciser ici quelques motifs qui nous conduiront à ne pas voter en faveur de la suppression de l'article 9. On peut effectivement, comme nos collègues socialistes, se demander ce que vient faire cet article dans un texte sur le droit du travail, lequel se retrouve ici dans l'orbite du droit fiscal. L'article 9 aurait donc les apparences d'un « cavalier » législatif, les dispositions modifiées ne pouvant l'être que par une loi de finances, puisqu'il s'agit ici d'articles issus de la seconde partie de la loi de finances pour 2017, dont l'examen n'a pas eu lieu au Sénat.

fiscale, mais un débat politique de fond sur le sens que l'on souhaite donner à notre système de prélèvements dits « obligatoires ». En effet, il est notamment question, depuis le début de la législature en cours, de procéder à quelques mutations de notre droit. La moindre n'est pas de réduire de manière assez sensible la taxation du capital et des patrimoines,, dans un premier temps, la et la sortie des revenus financiers de l'assiette de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement libératoire de 30 %, qui solderait l'affaire, autant pour les finances sociales que pour les finances de l'État. Comme les différentes contributions sociales actuelles atteignent 15,5 %, on imagine donc que la part restant au budget de l'État sera de 14,5 %, taux assez éloigné, éloigné, chacun en conviendra, des 45 % du taux d'imposition maximal du barème ! La réforme fiscale qui se dessine, en filigrane, derrière la mise en oeuvre de la retenue à la source, revient à solliciter de manière plus importante les couches modestes

par un impôt direct de plus en plus proportionnel, notamment le rapprochement de la CSG et de l'impôt sur le revenu et un allégement de fiscalité pour les revenus les plus aisés. collègues, la disparition du quotient familial inquiète assez peu les ménages fortunés, qui ont bien d'autres moyens de réduire la facture ! Voici pourquoi, en quelques mots, nous ne voterons pas cet amendement de suppression de l'article 9.

d'abord qu'il ne s'agit pas d'une disposition organique. Ensuite, nous avons tout à fait le droit de reporter la mesure ; c'est même la bonne gestion fiscale qui commande de prévenir dès maintenant, au coeur de l'été, après un débat présidentiel très important sur ce sujet notamment, que nous la reportons. En outre,

qui représente un danger tant pour le devenir des prélèvements fiscaux et sociaux que pour les citoyens, dont l'impôt personnel augmenterait à coup sûr. Il tend également à instituer un comité de suivi régional le CICE, pour s'assurer que les TPE et PME en bénéficient. Selon le droit actuel, lorsque le comité d'entreprise constate que le CICE n'est pas utilisé conformément à son objet, il peut demander des explications à l'employeur. Si l'employeur refuse de s'expliquer ou si l'utilisation non conforme du CICE est confirmée, le comité d'entreprise peut rédiger un rapport qu'il transmettra au comité de suivi régional du CICE. En l'état, le dispositif n'est pas suffisamment effectif. L'absence de sanctions peut décourager l'action des représentants du personnel. Quel

Les charges à payer au titre du CICE par le budget pour les remboursements de l'impôt sur les sociétés s'élevaient à 15,2 milliards d'euros en 2016, et le stock de créances était de 17,11 milliards d'euros à cette période, soit 17,11 milliards d'euros non consommés, mais qui devront être couverts dans les prochains budgets. Une augmentation de 5 milliards d'euros de crédits sera nécessaire en 2018.

mais ils ne mentionnent aucunement les Français de l'étranger. J'aimerais pourtant vous dire combien cette disposition suscite d'interrogations et d'inquiétudes parmi nos compatriotes expatriés et leurs élus, les conseillers

enfin, et tout particulièrement, parce que le crédit d'impôt pour éviter le double prélèvement pendant l'année de transition pourrait présenter de sérieuses difficultés. Nous souhaiterions

Cela s'est traduit par la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en 2010, alors que le secteur n'avait créé que 18 000 emplois sur les trois années précédentes. Une telle mesure semble donc aller dans le bon sens. J'espère que le Gouvernement inscrira le crédit d'impôt immédiat pour les particuliers-employeurs dans le prochain projet de loi

Notre amendement vise à supprimer l'article 2 de la loi dite El Khomri qui, vous vous en souvenez, avait inversé la hiérarchie des normes et permis de fixer des règles moins favorables aux salariés dans les domaines de la durée du travail, des repos et des congés payés. Depuis 2004, les réformes successives du code du travail ont étendu petit à petit les domaines dans lesquels les accords d'entreprise peuvent déroger aux accords de branche. Avec cet amendement, nous souhaitons rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur en droit du travail, afin de revenir sur les possibilités de déroger aux accords de branche par accord d'entreprise autrement que dans un sens plus favorable aux salariés. L'article 2 de la loi El Khomri a porté, nous le savons, un coup sévère aux droits des salariés, mais également aux petites entreprises, de sorte que

La loi El Khomri, qui a largement détricoté la durée légale du travail, ne suffit visiblement pas, car le Gouvernement souhaite encore aller plus loin avec ces ordonnances.

ou encore la modification du montant de l'indemnité de précarité. Le Gouvernement semble donc vouloir également mettre en concurrence les travailleurs entre eux en favorisant la baisse des salaires. comme nous l'avions dénoncé à l'époque, le gouvernement Valls a ouvert la voie dans laquelle l'actuelle majorité présidentielle s'engouffre aujourd'hui pour créer un code du travail au niveau de chaque entreprise. Notre amendement pose donc la question du choix de la société que nous voulons : une société du « chacun pour soi », où les droits des salariés dépendront du rapport de force dans l'entreprise, ou une société qui garantit des droits collectifs à tous les salariés, quelle que soit leur entreprise.

Personne ne demande plus à voter ?

les causes du chômage sont ailleurs. Il aurait fallu davantage s'attaquer à la modernisation de notre outil de production par des politiques industrielles volontaristes et à une meilleure répartition des richesses pour soutenir une relance économique, écologique et sociale.

de l'ordre public social. Or l'ordre public social n'est pas simplement protecteur de notre modèle social, il est aussi porteur de l'égalité républicaine.

il y aura plus de reculs que d'avancées. Il faut dire que les amendements du rapporteur, au nom de la commission des affaires sociales, y auront largement contribué. Je citerai pour exemple l'amendement COM-16 sur l'alinéa 12 et les dérogations concernant les entreprises de 11 à 50 salariés, ou l'amendement COM-17 explicitant le référendum d'initiative patronale. Si la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit quelques flexibilités, elle a aussi mis en place de réelles contreparties progressistes face à la baisse des risques existant pour les patrons des TPE-PME. Cette loi dite El Khomri a ainsi prévu le compte pénibilité, les congés spéciaux pour les événements familiaux, le droit des salariés dans le cadre des emplois saisonniers, le droit à la déconnexion, et

la suppression du motif économique pour les salariés refusant la modification de leur contrat de travail à la suite d'accords collectifs, la suppression des accords de maintien, l'inversion de la charge de la preuve et la réduction des délais de contestation, la suppression du mandatement, le référendum d'initiative patronale,

l'enrichissement de certains et la performance économique des entreprises tireraient tout le monde vers le haut. Il y aurait plus d'emplois, avec de meilleures rémunérations. C'est en gros

L'inversion de la hiérarchie des normes au profit d'une plus grande latitude de négociation au niveau de l'entreprise est indispensable pour que notre économie reparte en créant des emplois. Nous devons faire confiance aux partenaires sociaux : ils partagent un destin commun. de la discussion de la loi dite Macron, j'avais présenté un amendement appelant à modifier l'article 1 du code du travail pour permettre cette inversion de la

Madame la ministre, je profite de cette intervention pour vous dire notre étonnement devant votre refus de répondre, hier, à la quasi-totalité de nos observations et interpellations, qui démontraient sans ambiguïté les reculs qu'induit pour les salariés votre projet de loi.

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a publié un tableau détaillant les trois domaines d'application différenciée de la hiérarchie des normes. Des sujets qui relevaient de la loi, comme l'utilisation des contrats courts ou les CDI de chantier, pourront être mis en discussion au niveau de la branche. la primauté donnée à l'accord d'entreprise va délocaliser la négociation collective là où le salarié est le plus en situation de faiblesse. Le principe de « subsidiarité » dont vous parlez n'est là que pour brouiller les pistes. Il est en fait un principe de défaveur : c'est la possibilité donnée aux employeurs, éventuellement même en contournant les organisations syndicales, de remettre en cause des avantages garantis jusque-là par des conventions collectives. Nous en donnerons des exemples précis. précis. Vous proposez en fait l'adaptation des hommes aux besoins du marché de l'emploi. Quel progrès ! Au contraire, nous avons plutôt besoin de repenser le travail pour émanciper les hommes en créant des droits nouveaux pour protéger les travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.

licenciements. Vous vous trompez de voie, madame la ministre. Au lieu de faire un code du travail pour sécuriser les patrons des grandes entreprises, vous feriez mieux de faire un code du travail pour protéger les salariés et répondre aux défis du XXIsiècle.

axer mon propos sur l'article 1 du point de vue des travailleurs en situation de handicap. Alors que les entreprises de plus de vingt salariés sont dans l'obligation de recruter 6 % de travailleurs en situation de handicap, les chiffres sont accablants

Pire, ces travailleurs restent en moyenne 200 jours de plus sans emploi que les personnes n'étant pas en situation de handicap. Nous parlons tout de même ici d'une moyenne de 755 jours, soit plus de deux ans ! Au vu de la situation financière de l'AGEFIPH par rapport aux besoins réels, on peut légitimement s'interroger sur l'effectivité du versement obligatoire par les employeurs ne respectant pas leur obligation légale de recrutement. Si certains éléments extérieurs comme l'âge moyen

Crainte d'une mise en accessibilité coûteuse des locaux, crainte devant une adaptation nécessaire du poste de travail, appréhension face à une plus faible efficacité présumée des travailleurs en situation de handicap : les freins à l'insertion professionnelle sont encore nombreux. La situation est grave, alors que le handicap concerne plus de 12 12 millions de personnes dans le pays. Le projet que vous nous présentez va-t-il créer les conditions pour dépasser les difficultés que je viens de pointer, alors qu'il permettrait un nouvel affaiblissement des obligations des entreprises en rognant sur les prérogatives de la branche, pourtant plus protectrice, et surtout en capacité de raisonner à l'échelle de tout un secteur ? Comment ne pas voir que la primauté accordée à l'accord d'entreprise va permettre à des entreprises de s'exonérer de leurs obligations ? Parce que les préjugés sont encore forts, parce qu'un certain nombre d'employeurs craindront qu'une politique inclusive de leur part leur fasse prendre du retard sur leurs concurrents directs,

Aujourd'hui, un énième plan vient menacer les derniers emplois restants et l'équilibre de toute la plateforme chimique de Pont-de-Claix, qui a vu se succéder, depuis 1980, les plans de restructuration, les plans de sauvegarde, les plans de départ volontaire dans une pure stratégie financière laissant sur le carreau Au fil du dépècement de l'entreprise historique, Rhône-Poulenc, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, les conditions de travail des salariés se sont détériorées, alors qu'ils n'ont eu de cesse de défendre leurs emplois et la pérennité de leur site. La seule réponse que vous leur apportez est celle du MEDEF : hausse du temps de travail, baisse des rémunérations, souplesse des licenciements, suppression des indemnités sans moyen de recours. C'est la même solution que vous apportez d'ailleurs aux salariés de Schneider Electric, où tous les accords ont été annulés en application de la loi El Khomri, ou encore aux salariés de General Electric Hydro, auxquels la direction vient d'annoncer un plan social, avec la suppression de 345 emplois, c'est-à-dire la moitié des effectifs du site, ce qui signifie, à très court terme, l'arrêt de la conception, de la fabrication et de l'entretien des turbines pour les barrages EDF,

Des accords avaient pourtant été trouvés par M. Macron, alors ministre de l'économie de François Hollande pour non seulement créer des emplois, mais aussi assurer la pérennité du site. Votre texte est à l'image de ces accords passés : du vent, du bon vent dans les voiles du patronat pour lui permettre de gonfler ses profits, au détriment des salariés, pour qui ce vent est bien aigre. De plus, cela va à l'encontre des intérêts industriels et économiques de notre pays, ce que ni les salariés ni les parlementaires communistes ne peuvent l'accepter.

L'article 1 de ce texte vise à donner une place centrale à l'accord d'entreprise, et va donc renforcer le social dans notre pays. Jusqu'à présent, les domaines où l'accord d'entreprise pouvait déroger à l'accord de branche en fixant des règles moins favorables aux salariés étaient lissés et précisés. Le projet de loi d'habilitation prévoit d'inverser la règle en établissant la liste des domaines où l'accord de branche continue

demain, le renvoi au niveau de l'entreprise de la négociation sur la rémunération semble pouvoir autoriser les employeurs à négocier les primes d'ancienneté ou le treizièmemois,

La boîte de Pandore a été ouverte, permettant l'inversion de la hiérarchie et des normes et la suppression du principe de faveur, entraînant un social aggravé dans notre pays. Sous prétexte que la mondialisation de l'économie impose aux entreprises françaises d'être réactives,

Si l'idée forte retenue est celle de la primauté de l'accord d'entreprise, la branche est renforcée- je veux le souligner -dans un rôle essentiel de régulation des conditions de concurrence et de définition des garanties économiques et sociales. C'est vrai ! Je veux être plus précis

L'articulation est ainsi construite sur trois blocs de compétences, avec l'affirmation que les acteurs de l'entreprise ou de la branche sont suffisamment matures pour construire du droit applicable au sein de celle-ci. Cet article dessine le profil d'une entreprise où le principe de subordination n'est pas nié, mais où, à la culture des rapports de force et de l'affrontement conflictuel, se substituerait une culture du compromis résultant du diagnostic partagé, du dialogue, de la négociation, qui pourrait peut-être conduire, à terme, à la situation allemande de la codétermination. L'article 1 rouvre donc le débat sur l'inversion de la hiérarchie des normes. Il nous remémore, mes chers collègues, le long chemin parcouru depuis une ordonnance Auroux du 16 janvier 1982, prise par le gouvernement Mauroy II,

Lors de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications résultant d'un accord collectif, un point d'alerte porte sur le type de licenciement, ses modalités et le montant des indemnités de licenciement. Le point le plus sensible réside, à mes yeux, dans la situation des petites entreprises qui ne disposent pas de délégués syndicaux et pour lesquelles le système du mandatement ne fonctionne pas. La question centrale est celle de l'exclusivité syndicale dans la négociation d'entreprise. La remettre en cause serait franchir

Ainsi, l'article 1 jette les bases d'un droit nouveau, différent, se caractérisant par un équilibre entre, d'une part, la loi, qui continue de fixer les principes fondamentaux de l'ordre public- droits à la formation, à la protection chômage, égalité entre la femme et l'homme, interdiction des discriminations, mais aussi SMIC, durée légale du travail à 35 heures -et, d'autre part, des négociations de branche et d'entreprise qui fixent les règles communes et de proximité du monde du travail. Très bien

Il l'a fait avec le souci de favoriser le dialogue social à tous les niveaux par une meilleure articulation des conventions collectives au niveau national, conventions de branches et, surtout, accords d'entreprise, car c'est au sein de l'entreprise que les relations sociales se développent d'abord. J'adhère, pour ma part, pleinement aux lignes directrices adoptées par nos commissions compétentes. Je tiens à rendre un hommage appuyé à notre rapporteur, M. Alain Milon, et au rapporteur général de la commission des finances, M. Albéric de Montgolfier, pour leur excellent travail, en particulier sur l'article 1 tel qu'il nous est soumis, qui donne au débat un cadre sérieux et légitime. Il serait très regrettable que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'en tiennent aucun compte, se bornant à revenir purement et simplement au texte initial, comme c'est en ce moment le cas sur le texte « rétablissant la confiance dans l'action publique ». De plus, je voudrais attirer l'attention du Gouvernement sur la situation de nos compatriotes résidant à l'étranger qui vont subir de plein fouet les mesures diverses d'augmentation de la CSG ou de suppression de la réserve parlementaire, cette dernière contribuant à financer certains équipements nécessaires, en particulier pour l'amélioration de la vie scolaire et les Alliances françaises. Il nous a été dit que ce gouvernement souhaitait confier à de « hauts fonctionnaires » les décisions d'attribution, alors qu'ils n'ont pas une connaissance suffisante du terrain et des besoins spécifiques de chaque pays que les parlementaires, eux, connaissent parfaitement pour les visiter « physiquement » régulièrement. Enfin, il faudra que les gouvernements se souviennent, « hors des périodes électorales », que les Français résidant à l'étranger qui les ont élus sont des Français comme les autres et qu'ils ont droit à la même considération du Gouvernement que les Français de métropole et d'outre-mer.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, l'article 1 est bien le coeur de ce projet de loi d'habilitation dans la mesure où il réaffirme et précise la primauté des accords d'entreprise, mais aussi l'équilibre et l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Les principes, les dispositions d'ordre public demeurent du niveau de la loi. Un certain nombre de compétences restent du domaine exclusif de la branche, d'autres peuvent être déléguées aux entreprises dans le cadre d'accords de branche et la souplesse dérogatoire s'applique au niveau de l'entreprise. En tout état de cause, la branche demeure un niveau supplétif incontournable. Pour bien couvrir tout le champ des accords collectifs, il est nécessaire que la restructuration des branches professionnelles soit effective. À cet égard, j'exprimerai une petite nuance en termes de calendrier avec la position de la commission, car il me semble qu'un délai de dix-huit mois doit être suffisant pour la réorganisation des branches. En effet, dans beaucoup de domaines, nous préconisons plus de pragmatisme, plus de réactivité par la réduction des délais. Il n'y a pas de raison de ne pas demander cet effort aux branches professionnelles. Nous approuvons donc les orientations de cette loi et les inflexions adoptées par notre commission des affaires sociales sur cet article 1, en espérant, madame la ministre, que vous retiendrez l'essentiel des propositions constructives émises par la commission. L'une de ces dispositions, madame la ministre, constitue le marqueur essentiel de ce texte : celle qui doit permettre de multiplier les accords d'entreprise dans les PME et TPE. La loi du 8 août 2016, qui avait pour objectif d'encourager ces accords d'entreprise, introduisait dans les PME et TPE un dispositif de conclusion des accords qui allait à l'encontre même de cet objectif en imposant soit la présence d'un délégué syndical- or, il n'y en a que dans 4 % des entreprises de cette taille -, soit une procédure de mandatement, contrainte inadaptée si l'on veut obtenir des résultats significatifs en termes de nombre d'accords conclus. Je me félicite donc des dispositions différenciées pour les PME et TPE, en formulant cependant une remarque personnelle : pour définir des PME et TPE, nous ne pourrons pas effacer la notion de seuil, débat récurrent dans notre assemblée. Il me paraîtrait aujourd'hui raisonnable de remonter le seuil de 10 à 20 salariés, mais de conserver celui de 50 salariés, qui correspond à une définition européenne. Je veux souligner que la mise en place d'une instance unique de représentation du personnel est susceptible d'atténuer les préventions des chefs d'entreprises à franchir ledit seuil. La parole est à M. Martial Bourquin, Monsieur le président, permettez-moi de me joindre aux différentes congratulations exprimées par tous nos collègues sur l'ensemble des travées. Madame la ministre, mon intervention se fera sur le principe même des ordonnances. Quelle urgence y a-t-il à légiférer par ordonnances, à légiférer pour 18 millions de salariés et modifier le code du travail, qui doit être protecteur ? Quelle urgence ? J'ai vu que le Conseil d'État nous faisait part d'inquiétudes. Dans l'avis qu'il vous a remis, il constate en effet que le projet de loi contient un très grand nombre d'habilitations permettant au Gouvernement de prendre des ordonnances sur des sujets d'une portée et d'une complexité inégales. Il appelle l'attention du Gouvernement sur les conséquences d'un tel choix en termes de hiérarchie des priorités, de calendrier et de temps nécessaire à la préparation de ces différentes réformes. Alors, quelle est l'urgence ? J'essaie de comprendre, car il y en a certainement une,

plus d'une évaluation des conséquences économiques, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées

! Certains économistes nous disent pourtant que bien vivre avec une bonne santé au travail est certainement le meilleur facteur de productivité. Sur toutes ces questions,

Je souhaitais intervenir sur cet article pour rappeler que le contexte idéologique qui sous-tend le projet de loi que nous discutons aujourd'hui n'est pas neutre. J'irai même jusqu'à dire qu'il est discutable et discuté ! Je me permets ces rappels de base, après avoir écouté avec étonnement quelques affirmations sur ce texte et sur le code du travail, ces derniers jours. Madame la ministre, vous avez affirmé hier que notre droit du travail était devenu progressivement inadapté à l'économie de notre temps, non pas dans ses principes, mais dans ses détails. Peut-être cette inadaptation progressive est-elle due aux nombreuses réformes- dix-sept de 2000 à 2013, d'après Les Économistes atterrés ! -visant -visant à libéraliser le marché du travail ces dernières années, autant de réformes qui n'ont pourtant pas réussi à créer des emplois pérennes en nombre suffisant. Constatant les échecs passés, vous vous préparez à utiliser la même méthode : légiférer vite, sans même attendre le bilan complet des réformes du précédent quinquennat légiférer vite, et sans doute mal, pour éviter que nos concitoyens ne s'approprient un débat qui n'a pas été tranché lors de l'élection présidentielle ; légiférer vite, en utilisant des exemples européens bien peu convaincants. Ainsi, il est souvent de bon ton d'appeler la France à se réformer sur le modèle de l'Italie ou de l'Espagne, autant de pays où le taux de chômage est encore supérieur à celui de la France, malgré une démographie largement différente, mais il faut copier Renzi, il faut imiter Rajoy ! Aujourd'hui, madame la ministre, vous souhaitez légitimement soutenir la ligne défendue par le Président de la République réformons pendant que la cote de popularité est élevée, pendant la torpeur de l'été, pendant que l'ancien monde politique est encore tétanisé ! Mais il reste dans ce pays quelques millions de personnes qui estiment que cette philosophie de la dérégulation n'est pas pertinente socialement et qu'elle n'est pas efficace économiquement, parce qu'elle n'a pas fait la preuve de son efficacité ailleurs, parce que, en France, comme l'indique l'OCDE, les rigidités alléguées du marché du travail ne sont étayées ni en matière de licenciement individuel ni en matière de licenciement collectif, parce que ces dérégulations ont des effets pervers sur le travail des femmes, sur la précarisation de l'emploi, sur l'incitation des employeurs à toujours préférer la réduction des coûts à l'investissement. C'est pour ces raisons, sur la forme et sur le fond, que je m'opposerai à ce texte.

faveur : accepteriez-vous de partager une petite parcelle de la formidable ovation qui vous a été adressée avec tous nos collègues que nous ne reverrons plus, parce qu'ils sont touchés par cette loi absurde qui interdit le cumul des mandats ? La parole

qu'au sein d'une entreprise, quelle que soit sa taille, l'attention et la solidarité humaine et professionnelle sont bien aussi efficaces que les contraintes légales et financières pour faire place aux salariés avec handicap. Les outils existent, il faut savoir s'en saisir et c'est au coeur même de l'entreprise que cette conversion C'est par l'expérience collective, au plus près de la pratique, que l'on garantit la meilleure reconnaissance de la place des personnes handicapées et la défense de leurs droits de travailleurs. Nous saisissons l'occasion de cette loi d'habilitation à prendre par ordonnances des mesures pour le renforcement du dialogue social pour demander que le Gouvernement mène systématiquement des études d'impact des réformes envisagées sur l'emploi des personnes en situation de handicap et des proches aidants, tant en matière d'accès, d'évolution professionnelle que de maintien dans l'emploi, de façon à généraliser et rendre habituelle l'obligation de recrutement de 6 % de personnes handicapées dans les effectifs salariés, que l'entreprise soit publique ou privée.

Lors de la campagne présidentielle, le candidat Macron avait annoncé cette loi. Il avait annoncé qu'il la ferait débattre au Parlement et qu'elle serait appliquée par ordonnances.

! En même temps- pour employer une expression qui fait florès -, qui a peur de discuter dans une PME ? Pour ma part, je tiens le même discours dans la Drôme et à Paris.

Alors, madame la ministre, nous nous exprimerons dans ce débat avec des voix diverses, mais nous avons tous le même objectif, que la France se redresse

Pierre Gattaz disait qu'il faut donner la possibilité aux chefs d'entreprises de négocier le plus de choses directement avec les salariés. Il disait aussi que l'accord de branche ne doit primer que par exception.

les salariés sont une nouvelle fois la cible, sans qu'aucune évaluation de ces lois ait été réalisée, alors même que le président Macron vante l'évaluation des politiques publiques ! J'ai bataillé, avec l'ensemble de mon groupe, contre tous ces textes. Pourtant, chaque fois, vos prédécesseurs ne tarissaient pas d'éloges sur les mérites de ces nouvelles réformes. On nous assurait que, grâce à elles, le chômage allait enfin diminuer, que les entreprises allaient enfin pouvoir embaucher plus facilement ... Permettez-moi d'en douter, non seulement, quand je regarde l'état du pays, six ans plus tard, mais également parce que vous avez à nouveau besoin de prévoir une grande réforme qui poursuit et amplifie les attaques de la loi El Khomri, contre laquelle la rue a grondé durant des mois,

Pourtant, le texte parle pour vous : il y est indiqué noir sur blanc que le projet de loi entend donner à la négociation d'entreprise un rôle essentiel, et ce dans des domaines qui, jusqu'ici, relevaient de la branche ou de la loi.

L'idéologie néolibérale s'est attaquée au code du travail, dont on veut absolument faire un bouc émissaire, parce qu'il protège les salariés. Veillons donc à remettre les choses à l'endroit. Selon un rapport du FMI,

de l'impôt sur la propriété et d'une fiscalité plus redistributive. Je vous signale, mes chers collègues, que c'est absolument le contraire de ce que fait le Gouvernement, qui choisit de frapper les plus pauvres par la

Il n'y a pas de bouleversement de la hiérarchie des normes, car la loi reste évidemment supérieure à la négociation collective. Depuis 1982 et, surtout, depuis 2004 et la loi Travail de l'an dernier, le législateur donne à l'accord place centrale pour fixer les relations individuelles et collectives du travail. Beaucoup parlent d'un risque de concurrence déloyale au sein des branches, mais de nombreux garde-fous existent encore dans ce projet de loi D'une part, six thèmes relèvent déjà du monopole légal des accords de branche, comme les salaires minimaux, la classification ou l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En outre, la branche pourrait bientôt avoir le monopole de la fixation des règles en matière de gestion et de qualité de l'emploi, afin de définir un socle commun à l'utilisation des CDD, des contrats d'intérim et des CDI de chantier. D'autre part, sur les matières dans lesquelles un accord d'entreprise peut intervenir, il faut un accord entre les syndicats et l'employeur.

de mandat, ce texte ? -me semble déplacée. En effet, il vaut mieux faire de telles réformes en début de mandat et être tranquille par la suite pour faire en sorte que l'économie de notre pays puisse évoluer dans le bon sens et que le nombre de chômeurs puisse diminuer.

de l'article 1, je voudrais d'abord confirmer que, bien évidemment, la loi s'impose à tous. Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes en ce qui concerne la loi ; d'ailleurs, ce serait inconstitutionnel.

Or sur ce point, comme vous avez pu le constater, l'ensemble des organisations représentatives patronales et syndicales exprime plutôt un certain contentement sur l'équilibre qui a été trouvé

la mutualisation des financements paritaires, qu'il s'agisse du fonds de financement du paritarisme, des fonds d'information professionnels, des fonds de prévoyance, de la complémentaire santé et des compléments d'indemnité journalière.

Le deuxième bloc sera constitué de domaines pour lesquels nous considérons que la branche est compétente pour négocier. Ce sera à la branche de déterminer si ces

vote. Monsieur le président, je tenais à vous dire que les gentils mots que vous m'adressiez chaque fois que vous me rencontriez vont me manquer. En somme, vous allez quand même me manquer même me manquer ! Je voterai pour les amendements de suppression de l'article 1 de ce projet de loi, article dont la principale conséquence est le bouleversement profond de l'ordre public social français. Renverser la hiérarchie des normes, et donc favoriser une sorte de concurrence au sein de chaque branche, a des conséquences graves pour nos concitoyens. Nombre d'autres mesures constituent également un important recul pour les droits des salariés : l'inversion de la charge de la preuve et la fin du principe de faveur pour le salarié n'en sont que deux exemples. De surcroît, quelles que soient la pertinence de ce projet et l'urgence à intervenir pour « engager une réforme profonde du modèle social », nous ne pouvons que regretter, en tant que parlementaires, que le débat ne puisse avoir lieu au Parlement, par l'examen d'un projet de loi simple sur une question aussi complexe et importante, et qu'on ait plutôt recours à des ordonnances. Très bien ! L'ambition du président de notre « start-up nation » semble surtout être de faire adopter cette réforme pendant l'été, dans la torpeur du du mois d'août. Mais que l'on ne s'y trompe pas : il ne s'agit ici ni d'innover ni d'inventer le droit et la protection du travail pour les nouveaux statuts précaires, précaires, autoentrepreneurs, faux indépendants ou travailleurs des plateformes Uber et autres. Non, il s'agit surtout d'aligner le droit du travail à la baisse et d'offrir plus de précarité pour moins de droits. cela, en tant qu'écologiste, je ne me résigne pas !

La négociation suppose qu'il y ait un équilibre, que chacun soit dans une position qui lui permet, sans crainte et en toute sérénité, de négocier. Or cela ne sera pas le cas si le référendum est d'origine patronale. Vous indiquez également que l'accord collectif bénéficiera d'une présomption de légalité, ce qui signifie que le juge n'ira pas chercher ce qui, à l'intérieur de l'accord, peut être éventuellement illégal ; il faudra que le salarié apporte lui-même cette preuve, ce qu'il n'aura pas forcément la possibilité de faire.

pour ma part, aux auditions qui ont eu lieu sous l'autorité du président de la commission des affaires sociales, où nous avons entendu ces organisations.

faites le pari de la confiance envers les employeurs. Mais dans quel monde vivez-vous ? Nous sommes dans une société capitaliste.

pourtant que, lorsqu'une entreprise baisse les salaires et dégrade les conditions de travail, elle oblige par le mécanisme du capitalisme les autres à faire

mes chers collègues. L'ennui, c'est que le monde change : notre économie ne fonctionne plus comme au siècle dernier. Les échanges sont nombreux, rapides, internationaux ; les métiers évoluent, les marchés aussi.

et la loi vise à protéger les intérêts des plus modestes, c'est-à-dire des travailleurs les plus faibles, contre les excès de certains patrons qui n'ont pas encore compris le sens du dialogue social, celui de la solidarité et celui de la devise républicaine- liberté, égalité, fraternité.

L'endroit où l'on doit parler, c'est le Parlement, et ceux qui doivent parler, ce sont les parlementaires ! À partir du moment où vous nous proposez de régler un problème aussi important que celui du code du travail, c'est-à-dire le droit des salariés à la dignité dans leur travail et à leur épanouissement grâce au travail, vous n'avez pas le droit de vouloir légiférer par ordonnances, car vous privez le Parlement de son droit essentiel et les parlementaires de leur droit de base, à savoir parler et discuter de ce sujet. C'est pourquoi, madame la ministre, je ne voterai pas

Contre le chômage, la dérégulation n'a pas marché. C'est pour cela qu'il ne faut pas poursuivre dans cette direction. Pourquoi ces amendements de suppression ? Primauté de l'accord d'entreprise sur le contrat de travail et sur la question des branches, extension du contrat de chantier à d'autres secteurs que le BTP, niveau plancher et plafond des indemnités en cas de licenciement abusif, pouvoir de négociation de l'instance unique de représentation du personnel dans les entreprises de plus de cinquante salariés, modification du périmètre de l'appréciation du licenciement économique,

La messe est dite,

3 tend à renforcer considérablement la place des accords d'entreprise dans le droit social. En effet, il vise à définir de manière limitative les domaines dans lesquels les dérogations par des accords d'entreprise ne seront pas permises. Ainsi, tout domaine n'entrant pas dans cette définition pourra faire l'objet d'un accord

an. Sous prétexte de simplifier le code du travail et de renforcer les droits des travailleurs, cet alinéa revient en réalité sur le principe de faveur. Or il est déjà possible de négocier des accords au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, à condition qu'ils soient plus favorables aux salariés. Votre but, non pas de renforcer la négociation, laquelle est déjà possible, ou de la simplifier, mais bien de revenir sur les droits des salariés. Par ailleurs, une telle mesure ne ferait finalement que complexifier le droit du travail. En effet, c'est un peu comme si l'on envisageait un code de la route

quelques domaines qui demeurent du ressort de l'ordre public, voire de la branche, tout pourra se faire à la carte dans les entreprises. Et dans le cas où la branche continuerait à prédominer sur l'entreprise, cette dernière pourra encore déroger à la loi. Vous allez même jusqu'à considérer que les conditions de sécurité pourraient dépendre de l'entreprise, alors que, chaque année, plus de 600 000 accidents du travail sont déclarés,

qui est mise en place et la suppression du principe de faveur produiront des effets négatifs. Jusqu'à présent, sauf exception dûment prévue, les salariés, par la négociation collective à l'échelle de leur entreprise, ne pouvaient obtenir que des améliorations,

impossible de déroger aux accords de branche par un accord d'entreprise ou par une convention. Certes, les intentions du Gouvernement sont précisées, notamment dans le rapport de l'Assemblée nationale, mais la rédaction actuelle de l'alinéa 3 est encore beaucoup trop floue et laconique.

dans cette liste un domaine aussi important que la prévention de la pénibilité. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que la nouvelle articulation des normes soit dans tous les cas la plus explicite possible et qu'elle protège au maximum les salariés.

absence de délégués du personnel, élaboration d'un règlement intérieur ... Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet alinéa.

en exigeant que l'on se penche tout particulièrement sur le cas des petites entreprises dépourvues de représentants du personnel. Nous nous opposons à cet alinéa particulièrement révélateur de la philosophie générale du texte,

à faire référence à l'article L. 2211-1 du code du travail, qui prévoit que les dispositions relatives à la négociation collective s'appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

à la philosophie de l'amendement n° 23 rectifié, mais je me pose des questions sur le caractère opérationnel d'une telle précision. Il revient à la loi de fixer l'ordre public et le cadre juridique dans lequel les partenaires sociaux de la branche pourront négocier. À quel moment une stipulation d'un accord d'entreprise se transforme-t-elle en distorsion de concurrence la commission a émis un avis défavorable

Il faut achever la dynamique portée par la loi Travail, qui vise à donner plus de place aux accords d'entreprise dans le code du travail. La commission émet donc un avis défavorable sur ces

pourrait aboutir à ce que la question de la pénibilité fasse partie non plus des thèmes relevant du premier bloc, celui du monopole légal des accords de branche, mais du deuxième bloc, celui des clauses verrouillées sur décision de la branche. En outre, la rédaction proposée alourdirait le texte, alors même qu'au moins cinq des six thèmes actuels devraient être repris par l'ordonnance. La commission a également émis un avis défavorable sur l'amendement n° 2 rectifié

des conventions de revitalisation. Il vaudrait mieux agir concrètement dans ce sens, plutôt que de réduire les protections des salariés.

Il me semble qu'il y a dans le projet de loi d'habilitation une sorte d'incohérence.

vote. Je ferai une proposition constructive. Dominique Watrin a fait allusion à un rapport extrêmement passionnant qui vient d'être adopté par le Conseil économique, social et environnemental sur le financement des PME

Cet amendement vise à sauvegarder la nécessaire équité entre les entreprises qui sont capables de signer des accords d'entreprise et celles qui sont dans l'incapacité de le faire. À partir du moment où le Gouvernement accorde une plus grande latitude aux accords d'entreprise, cet amendement vise à prévoir que dans les entreprises employant moins de onze salariés et dans celles employant moins de cinquante salariés dépourvues de représentant du personnel, le chef d'entreprise puisse déroger à l'accord de branche. Il s'agit de prévoir la souplesse suffisante dans l'entreprise en fonction de son activité et de sa situation. Ce faisant, cet amendement tend à refléter le dialogue social informel qui se tient quotidiennement dans les plus petites entreprises, dans lesquelles le chef d'entreprise est de fait proche de ses salariés, car ils partagent un même cadre de travail et un même vécu du métier. Les artisans, notamment, et les TPE attendent une telle possibilité de dérogation avec impatience. l'avis de la commission ? L'alinéa 4 de l'article 1 vise, à terme, à obliger les accords de branche à prévoir quelles sont les stipulations qui ne s'appliquent pas aux petites entreprises et à en adapter d'autres pour tenir compte des spécificités de ces entreprises, qui constituent, nous le savons tous, l'immense majorité de notre tissu économique. Nous avons déjà mis l'accent

par accord de branche, dans les entreprises employant moins de onze salariés et dans celles qui emploient moins de cinquante salariés, mais qui sont dépourvues d'institutions représentatives du personnel. Pour mémoire, l'article 63 ou loi Travail, a autorisé l'employeur, à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, à appliquer un accord type prévu dans un accord de branche, au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé les délégués du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. Cet amendement est donc plus précis et plus ambitieux que le projet de loi actuel. À titre personnel, je comprends parfaitement les motivations de notre collègue Philippe Mouiller et je rappelle que le Sénat avait déjà, l'an dernier, lors de l'examen de la loi Travail, souhaité conditionner l'extension d'un accord de branche à l'existence d'accords types au profit des petites entreprises. En tout état de cause, je souhaite savoir où en sont les négociations avec les partenaires sociaux sur ce point. La commission se rangera à l'avis du Gouvernement.

Il s'agit, notamment, de mettre en évidence le fait que des postes de travail puissent être amenés à disparaître et que les salariés jusqu'ici occupés à ces fonctions ne pourront plus suivre leur parcours professionnel.

La simple lecture des articles du code du travail évoqués dans cet alinéa se passe de commentaire. Comme cela concerne des situations légèrement différentes, les procédures qui ont pu être prévues dans ce cadre le sont tout autant. Plutôt que de jouer la mélodie du bonheur ou la cantate du progrès, on nous propose ici d'écrire la partition, en mode mineur et plutôt sinistre d'ailleurs, de la rengaine du licenciement pour motif personnel. Il n'aura échappé à personne que celui-ci s'avère moins protecteur des droits du salarié que le licenciement économique C'est sans doute ce que d'aucuns appellent « rendre effectifs des droits sociaux », puisqu'il s'agira probablement de les réduire. Évidemment, quelques fins esprits ne manqueront pas de nous indiquer que de telles procédures ne pourront être mises en oeuvre que dans le cadre d'accords négociés, fruits d'un dialogue social sans cesse amélioré et renouvelé, mené au plus près du terrain, jusqu'à l'entreprise elle-même. Néanmoins, le dialogue nécessite que l'ensemble des tenants et aboutissants de l'affaire soient dans l'esprit de chacune des parties. Or, comme dans les entreprises nous sommes plutôt habitués à une certaine violence des échanges, il est juste à craindre qu'en ce domaine, comme en bien d'autres, l'accord « au plus près du terrain » ne soit pas en faveur des salariés. C'est la raison pour

droit au contrat de sécurisation professionnelle qui permet une meilleure indemnisation du chômage. Il s'agit d'une mesure de justice sociale lors d'un licenciement. Toutefois, l'ordonnance prévoit ici de modifier le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat issues d'un accord collectif, notamment d'un accord d'aménagement du temps de travail, d'un accord de maintien dans l'emploi ou d'un accord pour le développement de l'emploi, connus sous le nom d'« accords de compétitivité ». Or notre crainte est que cette simplification ne se fasse au détriment du travailleur : celui-ci pourrait alors subir un licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors qu'il refuse de se plier aux exigences du dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire à une baisse de son salaire, à une augmentation du temps de travail ou autre. C'est la question de l'équilibre du contrat qui est ainsi posée. Il faut rappeler ce que signifie l'abandon du motif économique : l'employeur pourrait se défaire de son obligation de reclassement, priver le salarié de tout contrat de sécurisation professionnelle ou de congé de reclassement et ramener son allocation chômage de 75 % de sa rémunération brute mensuelle, taux applicable en cas de licenciement pour motif économique, à 57 % seulement. Le contrat est censé représenter un équilibre : il est négocié lors de l'embauche, avec un nombre d'heures prévues, un salaire ... Bref, comme tout contrat, il offre une sécurité juridique. Cet alinéa tend à renforcer l'imprévisibilité

l'amendement du Gouvernement,

La suppression des accords de maintien dans l'emploi ne se justifie pas. L'objectif est différent, les accords de préservation et de développement de l'emploi, ou APDE, étant déconnectés des difficultés de l'entreprise et liés à de simples ajustements de l'organisation de l'entreprise à des variations d'activités, d'investissement ou de changement de conjoncture. De plus, les clauses de l'accord de maintien de l'emploi ne se substituent pas de plein droit aux clauses contraires des contrats de travail sans l'accord des salariés. Les licenciements éventuels reposent alors sur un motif économique.

pour les licenciements des salariés qui refusent l'application d'un accord de flexisécurité. Par ailleurs, notre rédaction écarte l'application des règles relatives à un plan de sauvegarde de l'emploi pour ce type de licenciement,

donc un licenciement, comme le législateur l'a prévu pour les APDE. L'employeur devrait donc, selon la commission, suivre une procédure spécifique unique et proposer aux salariés concernés un dispositif d'accompagnement lui aussi unique, présentant les mêmes garanties que le contrat de sécurisation professionnelle, actuellement réservé aux salariés licenciés pour motif économique. J'en viens aux amendements en discussion commune. Il

un soutien du Sénat à ces accords, dont nous souhaitons la disparition dans un souci de simplification juridique et d'allègement du code du travail. C'est pourquoi nous avons souhaité supprimé la référence à cet accord,

pendant la discussion générale, nous, sénateurs, avons pu nous forger nos propres convictions ces dernières années ; nous avons le droit, je dirais même le devoir, d'encadrer un projet de loi d'habilitation lorsqu'il s'agit de sujets aussi structurants. Je vous Je vous rassure, même en prévoyant un motif spécifique au licenciement, les partenaires sociaux auront encore beaucoup de grains à moudre. Il leur faudra en effet définir précisément la procédure du licenciement, qui sera distincte de celles applicables pour motif économique ou personnel, et créer un nouveau dispositif d'accompagnement transversal, sur le modèle de la convention de sécurisation professionnelle. La commission émet donc un avis défavorable sur

Or un accord d'entreprise peut concerner des sujets très sensibles, comme le travail de nuit ou l'annualisation des horaires de travail ; il ne doit pas jouir d'une telle présomption.

ni les temps de repos obligatoires. Or on sait à quel point ces éléments sont importants pour la sécurité des salariés, au-delà même de leurs conditions de vie.

Les alinéas 6 à 8 de l'article 1 tendent à rendre plus difficile la contestation des accords collectifs en agissant à la fois sur la charge de la preuve, les délais de contestation et les conséquences de l'annulation d'un accord. Le respect des droits fondamentaux des travailleurs se trouvera donc moins bien garanti qu'aujourd'hui. Comme le projet de loi entend renvoyer à la négociation d'entreprise une large partie des normes sociales, ces dispositions vont déséquilibrer les relations entre employeurs et salariés, en entravant la mise en cause d'accords qui seraient contraires à la loi. Nous proposons donc de supprimer les alinéas 6 à 8.

à limiter le contrôle du juge sur les accords collectifs en inversant la charge de la preuve, en réduisant les délais de contestation d'un accord. Preuve en est, s'il en était besoin, que vous ne faites pas confiance au juge prud'homal, Alors que ce projet de loi entend renvoyer à la négociation d'entreprise l'édiction de règles essentielles des normes sociales, ces dispositions visent uniquement à rassurer les employeurs, en rendant de plus en plus difficile la contestation d'accords qui seraient contraires à la loi. Sous prétexte de sécuriser l'application des accords collectifs, il faudrait réduire le délai pour dénoncer une disposition conventionnelle défavorable ou encore permettre au juge de moduler dans

Les revirements de jurisprudence et la rétroactivité des décisions du juge ont eu des conséquences lourdes pour les entreprises, comme lors de l'annulation de l'accord Syntec en 2013, qui permettait à 544 000 cadres de réclamer une revalorisation de leurs salaires. Jusqu'à maintenant, les droits des salariés ont toujours été pris en compte par le juge, contrairement à l'impact économique pour les entreprises. Or les décisions du juge peuvent placer ces dernières dans des situations financièrement dramatiques, qui dégradent leur trésorerie, dissuadent toute embauche et, finalement, se retournent contre l'ensemble des salariés. Il est donc essentiel de rappeler l'objectif de sécurité juridique visé par cette possibilité, pour le juge, de moduler dans le temps les effets de ses décisions. Les deux amendements suivants sont

triennale. Désormais, chacun fera comme il voudra ! Il y a fort à parier que certains employeurs ne s'embarrasseront pas avec ce qu'ils considéraient comme des contraintes inutiles et évidemment intolérables ... Il est vrai que les négociations sur les salaires et l'égalité professionnelle ne semblent pas si importantes

de convaincre nos collègues, ainsi que le Gouvernement. L'examen de ces dispositions, il y a deux ans à peine, avait permis de trouver un équilibre entre la nécessaire dynamisation du dialogue social et la préservation des prérogatives des instances de dialogue, lesquelles assurent une expression collective des salariés. À titre d'exemple, la périodicité des négociations annuelles obligatoires sur les salaires ou l'égalité professionnelle peut être adaptée par accord, la seule restriction étant que ces négociations doivent avoir lieu au moins tous les trois ans. Rouvrir ce chantier, alors que la réforme vient à peine d'entrer en vigueur, ne nous paraît pas opportun. Ce serait même une source d'instabilité juridique pour les entreprises. Or cette instabilité,

la formulation est vague, pourrait permettre à chaque entreprise d'adapter par accord la périodicité et le contenu des négociations annuelles obligatoires et des consultations, au-delà

S'inscrivant dans la logique de simplification de la loi du 17 août 2015, l'alinéa 9 pourra permettre à l'accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, aujourd'hui peser sur les entreprises du fait qu'elles sont insuffisamment coordonnées ou adaptées à la réalité de la progression du dialogue social. Il est utile que l'objectif de rationalisation soit clairement affiché pour garantir l'efficacité d'une telle mesure.

surtout en cas d'annulation par le juge, compte tenu des effets rétroactifs de cette décision sur les salariés et les employeurs. On ne peut pas encourager le développement des accords d'entreprise sans se soucier de leur sécurité juridique. Il est en effet essentiel de permettre au juge judiciaire, sur le modèle du juge administratif, de moduler les effets de ses décisions dans le temps, afin de permettre aux partenaires sociaux de conclure un nouvel accord ou un avenant qui purge les irrégularités décelées par le juge. L'avis de la commission est donc défavorable. identiques n 71 rectifié et 93, la commission n'est pas opposée à un aménagement de la charge de la preuve en matière de contestation des accords collectifs. Le Conseil d'État a, dans son avis, validé le principe de cette réforme, qui consiste à revenir au droit commun : c'est celui qui conteste un acte juridique qui doit apporter la preuve qu'il n'est pas qu'il n'est pas conforme au cadre légal. Il s'agit ainsi de tirer les conséquences d'une nouvelle jurisprudence de la Cour de la cassation, qui donne plus de poids aux accords collectifs.

de lutter contre l'insécurité juridique liée à l'annulation d'un accord collectif. Un délai de cinq ans pour attaquer directement un accord collectif en action en nullité paraît

rectifié vise à compléter l'habilitation sur la modulation des décisions du juge, en reprenant la rédaction d'un amendement que le Sénat avait adopté l'an dernier lors de l'examen de la loi Travail ; je rappelle à cet égard que c'est sans doute

Nombre d'employeurs et de salariés peinent d'ailleurs à suivre le rythme des réformes. Le sujet des négociations collectives a été revu en profondeur par la loi Rebsamen de 2015, tandis que la base de données unique existe effectivement depuis la loi du 14 juin 2013 Je n'ai pas souhaité supprimer cette habilitation en commission, en espérant que les modifications proposées par ordonnance seront partagées par les partenaires sociaux et ne remettront pas en cause l'équilibre des dispositions actuelles. L'avis de la commission est donc défavorable.

obligatoires dans les entreprises, la loi Rebsamen du 17 août 2015 a opéré une rationalisation autour de trois blocs. De fait, en application de l'article L. 2242-1 dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager chaque année deux négociations : l'une sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; l'autre sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur doit engager tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. La loi a en outre offert aux partenaires sociaux la possibilité d'adapter, par accord majoritaire, la périodicité des négociations obligatoires, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

décider de moduler les effets de sa décision dans le temps. Cette possibilité est pourtant rarement appliquée. La codification de ce principe serait donc utile, dans un souci de bonne intelligibilité de la norme, et pour laisser des marges d'appréciation au juge.